La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d'orientation des mobilités.

Par cohérence avec notre amendement n° 112, nous souhaitons que l'exigence de report modal repose également sur la définition d'un cadre social et fiscal qui permette d'en finir

Depuis des décennies, tout est mis en oeuvre pour favoriser à outrance le transport routier. Non seulement celui-ci ne s'acquitte pas du prix normal, mais, en plus, il est subventionné : exonération partielle de taxes pétrolières, abaissement de la taxe à l'essieu, tarifs des péages autoroutiers sans rapport avec l'usure causée par la circulation des camions, allégement des charges sociales, recours aux travailleurs détachés ... On le voit bien, tout a été fait pour faciliter le recours aux camions. Ainsi, selon la direction générale des douanes et droits indirects, le différentiel de taxation entre l'essence et le gazole entraîne une perte de recettes fiscales qui s'élevait en 2011, tous utilisateurs confondus, à 6,9 milliards

ferroviaire, d'autant plus que le président Rousset a toujours refusé de financer les infrastructures routières. Malgré cela, malgré les 1,4 milliard d'euros investis par le conseil régional, nos trains accusent deux fois plus de retards, du fait de la défaillance des infrastructures. C'est pourquoi je demande que nous puissions mettre en oeuvre un pacte ferroviaire régional. Il nous faut un plan ambitieux pour les lignes du quotidien. Comment peut-on exclure de toute solidarité nationale des lignes ferroviaires comme Bordeaux-Nantes, Limoges-Bordeaux ou même Limoges-Poitiers ? Ce sont des infrastructures structurantes pour notre pays

parole est à Mme la ministre. Le rapport annexé prévoit, d'une part, de renforcer la connaissance, l'entretien et la sécurité des ouvrages d'art, et, d'autre part, un accompagnement de l'État concernant le patrimoine des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cet accompagnement

par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le Cérema, qui anime des conférences techniques interdépartementales. Ces dispositifs seront consolidés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui aura vocation à appuyer les collectivités territoriales en matière d'ingénierie. Par ailleurs, en tant que gestionnaires routiers, les différentes collectivités disposent de la libre administration de leurs équipements, y compris en termes de choix de priorités et de politiques et de niveaux d'investissement, sans intervention de l'État. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de supprimer l'alinéa 30 du rapport

la réparation de ces ouvrages, qui présentent aujourd'hui de forts risques en termes de sécurité, mal connus. Il est difficile d'évoquer l'entretien et la modernisation des infrastructures sans aborder cette question très importante. Notre commission mène d'ailleurs actuellement un travail d'information sur ce sujet,

Cela n'est pas suffisant pour garantir la sécurité de près de 11 412 kilomètres de voirie et de 12 000 ouvrages d'art. Comme l'a rappelé le président de la commission, Hervé Maurey, le réseau routier connaît une dégradation continue depuis plusieurs années. Alors que plus de 85 % des chaussées étaient dans un état correct entre 2010 et 2012, ce taux est tombé à 83

à l'Afitf n'a été ni remplacée ni compensée, alors même qu'elle avait le mérite d'établir un lien entre l'utilisation de la voirie et la redevance. Dès lors, il est impératif d'enrayer dès à présent la baisse des crédits affectés à l'exploitation et à l'entretien de ce réseau routier. En effet, outre le risque d'atteinte au patrimoine, le défaut d'entretien des routes est un facteur déterminant d'accidents. Dans 40 % des accidents mortels, l'état des infrastructures est en cause. Comme le souligne le rapport réalisé l'été dernier par deux bureaux d'études suisses et remis au ministère des transports quelques jours après le drame de Gênes, « sans changement de politique majeur sur les infrastructures dans les prochaines années, plus de 60 % des chaussées seront très dégradées d'ici à 2037 ». Enfin, l'exemple du réseau ferroviaire devrait nous alerter : c'est un manque d'investissements dans l'entretien et la régénération du réseau qui explique son état dégradé. Quel est l'avis de la commission Même si elle déplore elle aussi l'insuffisance des moyens, la commission a fait le choix de ne pas augmenter les montants prévus par la trajectoire d'investissements dans les infrastructures, afin de privilégier la crédibilité de cette programmation.

sous-investissement chronique de l'État dans les infrastructures routières a pour conséquence l'implication de plus en plus fréquente des collectivités

Cette tendance lourde étant appelée à perdurer, le présent amendement vise à augmenter les crédits des contrats de plan État-région dans le scénario n°

En effet, dans son rapport, le Conseil d'orientation des infrastructures, ou COI, a confirmé que l'état de dégradation avancée du réseau fluvial nécessitait un sévère rattrapage, après des décennies de sous-investissement. Plus précisément, le COI estime que, pour maintenir la fonction de navigation sur l'essentiel du réseau, un budget de 245 millions d'euros par an serait nécessaire pendant dix ans-

termes, une part importante du réseau devra être fermée à la navigation, ce qui privera de nombreux territoires d'une desserte fluviale pour le transport comme le tourisme. À l'heure de l'urgence climatique, il est nécessaire de conserver l'intégralité d'un réseau qui garantit des prestations de transport trois à quatre fois moins émettrices de gaz à effet de serre que le transport routier

cette année, pour une livraison en 2023. Cet amendement est en tout point conforme à la volonté exprimée à de nombreuses reprises par toutes les collectivités des territoires concernés- départements, communautés d'agglomération et de communes, communes -, ainsi que par les forces économiques des différents départements. Il tend à exprimer les besoins des usagers. Ses dispositions du saut qualitatif nécessaire, en deçà duquel l'attractivité des dix départements directement concernés resterait insuffisante et ne permettrait pas le rééquilibrage des territoires que nous souhaitons tous. L'amendement

. Lorsque des lignes structurantes comme les trains d'équilibre du territoire, les TET, font l'objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures, l'État peut mener ces opérations de manière concomitante,

un programme de régénération des infrastructures, un renouvellement du matériel roulant et un programme de modernisation des infrastructures. Il paraît pertinent, tant au niveau budgétaire pour l'État et les régions participantes dans le cadre des contrats de plan État-région qu'au niveau de l'efficience des travaux et des perturbations entraînées par ceux-ci pour les usagers, que les phases de régénération et de modernisation des infrastructures aient lieu concomitamment. De plus, les travaux de modernisation ont pour objet, dans le cadre du Paris-Clermont-Ferrand, de permettre une réduction notable du temps de trajet. C'est l'un des objectifs essentiels de ces travaux, dont le résultat sera directement ressenti par les usagers. Il n'en est que plus nécessaire d'effectuer les travaux de manière concomitante.

Cet amendement est très attendu par les élus locaux, les usagers et les acteurs économiques concernés par les lignes d'équilibre du territoire, notamment la ligne Paris-Clermont-Ferrand, que je connais plus particulièrement et dont le temps de parcours, je le rappelle, s'est détérioré en trente Nous savons tous que la modernisation des trains d'équilibre du territoire constitue un élément stratégique majeur de l'aménagement du territoire. Les sénateurs comme le Gouvernement semblent aujourd'hui reconnaître cette nécessité. Ces lignes structurantes maillent et désenclavent les territoires, rapprochent les populations et constituent une alternative à la voiture et à l'avion, moyens de transport gourmands en énergies fossiles Pour les trains Intercités, on distingue trois phases de travaux : la régénération des voies, le renouvellement des rames et la modernisation du matériel roulant.

Ces amendements visent à prévoir que les travaux de régénération et de modernisation de ces infrastructures peuvent être menés de manière concomitante. Leurs auteurs font référence aux trains d'équilibre du territoire Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Toulouse. Ces projets sont phasés par un schéma directeur : il y a tout d'abord un programme de régénération des infrastructures, puis un renouvellement du matériel roulant, enfin une modernisation. La première phase et la deuxième phase devraient être menées concomitamment, selon les auteurs des amendements. Je comprends l'intention d'accélérer les travaux et de réduire les dépenses, mais je ne crois pas, comme je l'ai indiqué en commission, qu'il y ait aujourd'hui un obstacle à les réaliser concomitamment.

concomitamment. Je ne suis pas convaincue qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi, étant entendu qu'il n'y a pas de concurrence pour les moyens

J'aimerais juste citer l'exemple de l'Autriche, qui est pionnière avec son réseau de nuit transportant 1,4 million de passagers : on estime que 12 000 vols

qui ne bénéficient pas d'offres de rechange. J'ai également annoncé que nous allions investir 30 millions d'euros dans la modernisation du matériel. À plus long terme, ce matériel devra être renouvelé.

mais aussi le développement des liaisons tram-train inter-urbaines. Le transport par câbles peut être développé et favorisé dans les déplacements intra-urbains en complément des métros et bus, permettant ainsi de désengorger ces transports ou de créer de nouvelles lignes à moindre coût. De plus, ce mode de transport non carboné réduirait fortement la pollution des grandes villes. En montagne, il rendrait plus attractifs et efficaces les espaces valléens. Le développement du transport par câbles et des ascenseurs valléens est donc indispensable pour l'économie touristique de nos territoires, afin de désengorger l'accès aux stations lors des « migrations hivernales », mais aussi de faciliter et décarboner le transport au quotidien des habitants. Par ailleurs, développer la mobilité par liaison tram-train, lorsque celle-ci est possible, permettrait le désenclavement des territoires des transports décarbonés. Cela répond à un double enjeu d'attractivité des territoires et de réduction de pollution. Favoriser les transports décarbonés à un coût abordable pour l'usager, grâce aux transports guidés, tel est l'objet de cet amendement.

madame la ministre,

? Le Gouvernement s'est engagé à maintenir huit lignes dans le périmètre des trains d'équilibre du territoire, six lignes de jour et deux de nuit, étant entendu que dix-neuf

par l'opérateur public, et que cette offre revienne au goût du jour.

à la dégradation de la desserte de la région Normandie, qui, depuis les années 1970, est l'une des seules à avoir vu ses temps de trajet vers Paris augmenter. Or, sa mise en place ne cesse d'être reportée, et les transformations revues à la baisse. La description ici faite semble entériner un tel renoncement, puisque le découpage proposé et le phasage des différentes sections dans leur réalisation renvoient la partie proprement normande du projet à une date inconnue et lointaine. Alors que la date de lancement des enquêtes publiques pour la section Paris-Mantes est fixée à la période 2023-2027, aucune date n'est précisée pour la section Rouen-Barentin, sans même parler de la réalisation des travaux, qui est ainsi renvoyée à un futur très lointain. Il en va de même pour la section dénommée « Y de l'Eure », dont la réalisation a déjà été reportée au-delà de 2037. Le rapport annexé au présent texte ne se concentre finalement que sur la réalisation de la section Paris-Mantes, laissant de côté le reste de cette ligne pourtant censée traverser la Normandie jusqu'à Yvetot. La construction de la seconde gare de Rouen et celle de la traversée sous-fluviale qui doit l'accompagner sont ainsi négligées, alors même qu'elles constituent les mesures les plus efficaces pour soulager le noeud ferroviaire rouennais en situation de saturation. La perspective est d'autant plus surprenante

desserte ferroviaire du port du Havre, une avancée importante va être réalisée avec la mise en service, en 2020, de la liaison Serqueux-Gisors.

Or le Président de la République, au cours d'une réunion organisée dans la Drôme en début d'année dans le cadre du Grand Débat, est intervenu sur ce sujet.

parmi les grands projets d'infrastructures entrant dans le champ de programmation des investissements prévus à l'article 44. Ce projet, dont on parle depuis très longtemps, et même depuis des décennies, a reçu l'aval de plusieurs gouvernements jusqu'à aujourd'hui.

45 demeure nécessaire aujourd'hui pour désenclaver Saint-Étienne et sa région.

la réalisation de ce projet autoroutier : à la fois l'amélioration de l'autoroute A 47 et, surtout, le renforcement de la liaison ferroviaire Lyon-Saint-Étienne. Ces éléments figurant dans l'exposé des motifs, je propose, par

et, en même temps, le réaliser. À un moment, il faut bien prendre une décision, et c'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. Mme la ministre l'a rappelé : le contournement ouest de Lyon ne se fera pas.

là où « le fer croise le fer ». Dans une loi sur les mobilités, une loi du XXI siècle, l'intermodalité doit être une évidence et s'imposer.

Dans le rapport annexé sont pointés des programmes d'investissements prioritaires et la nécessité de remédier à la saturation des noeuds ferroviaires dans les grands pôles urbains. En clair, il s'agit d'améliorer les transports quotidiens en doublant la part du transport ferroviaire et en améliorant l'usage des transports déjà existants. En Île-de-France, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré doivent être approfondis, le but étant de remédier à la congestion des réseaux et à la dégradation des conditions d'usage des transports collectifs, tels que le métro, le tram ou le RER. À ce propos, je vais prendre quelques secondes pour parler

La section des accès français au Lyon-Turin a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2013. Celle-ci vise à accompagner le développement du fret ferroviaire en permettant de mener une politique forte et visible de report modal, tout en contribuant à la desserte des grandes agglomérations du sillon alpin Les réflexions doivent se poursuivre. Il s'agit de déterminer une programmation pertinente, afin de faire face dans la durée à l'accroissement des trafics, d'ici à l'ouverture de la section transfrontalière, prévue à l'horizon 2030, en mettant en service de façon échelonnée les tronçons nouveaux selon l'itinéraire Bas-Dauphiné, puis jusqu'en Maurienne. Parallèlement, un observatoire des trafics et des capacités des itinéraires

du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise et du noeud ferroviaire lyonnais. Ce projet de loi doit inclure les dispositions permettant de maintenir la dynamique globale de ce projet écologique et géostratégique dans le respect des engagements internationaux de la France.

Madame la ministre,

la capacité de ces derniers à coopérer et à se développer durablement de façon complémentaire et mutuellement bénéfique. Ce postulat se vérifie sur le terrain, quand les liaisons routières entre une métropole et les villes moyennes qui l'entourent sont performantes, qu'il s'agisse d'autoroutes ou de routes à 2x2 voies.,

affectées. Le développement induit par la métropole se fait alors en tache d'huile. Cette situation peut provoquer des difficultés de croissance pour les territoires qui l'accueillent et des difficultés de décroissance pour ceux qui en sont privés. De leur côté, les villes moyennes concernées ne peuvent pas jouer le rôle moteur qui doit être le leur dans leurs zones géographiques d'influence, espaces englobant les bourgs centres avec lesquels et au profit desquels elles sont en relations.

Pour ces raisons, et au nom de l'intérêt général, l'État doit engager et terminer le plus rapidement possible ces chantiers routiers à fort enjeu de développement territorial. Quel est l'avis de la commission

: La parole est à M. Éric Gold. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les aménagements qui doivent nécessairement être mis en oeuvre sur la portion lozérienne de la route nationale 88, pour engager le désenclavement de ce département hyper-rural.

entre l'A 75 et Langogne, l'ensemble des élus du territoire se sont entendus sur un objectif cible d'une mise à 2x2 voies sur la totalité de l'itinéraire, mais avec une définition de tronçons prioritaires acceptables financièrement et en adéquation avec les contraintes budgétaires de l'État. Pour le reste de l'itinéraire, des aménagements ponctuels sont envisageables, à condition qu'ils permettent à terme d'atteindre l'objectif cible d'une mise en 2x2 voies sur le tronçon lozérien de la RN 88.

ni de 2x2 voies, et encore moins d'infrastructures ferroviaires. Je ne vous en parlerai pas, tout simplement parce que le département que j'ai l'honneur de représenter ici ne possède aucun

: cette mesure permettrait aux élus et aux citoyens d'avoir connaissance des différents projets pour lesquels l'État s'est engagé.

et des territoires ruraux, il est prévu que l'État porte un programme d'une vingtaine d'itinéraires routiers au sein des CPER, pour un montant total d'un milliard d'euros sur dix ans. Ces projets visant à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national correspondent à des opérations concrètes sur les itinéraires existants, comme des déviations courtes, des aménagements de carrefours, etc. il est précisé également que ce programme prioritaire ne se fera pas au détriment de l'avancement des autres projets contractualisés dans les CPER. Or les CPER actuels portent sur la période 2015-2020. Il faudrait donc modifier la loi dès l'année prochaine pour tenir compte des nouveaux CPER. En outre, la liste de ces projets, qui est accessible, devrait également être actualisée dans la loi chaque fois qu'une modification serait apportée à chaque contrat, ce qui ôterait

de réaliser les contrats de plan sur lesquels l'État est engagé. S'agissant du rythme, je ne peux pas vous dire que cela se fait à une vitesse exagérée, mais notre ambition est bien de terminer ces contrats de plan

Des axes structurants et accidentogènes restent en attente d'une amélioration des conditions de circulation. Il est nécessaire d'ajouter ce critère pour déterminer les projets routiers inclus dans les contrats de plan État-région, afin d'assurer une meilleure sécurité routière.

Ni la programmation ni la loi n'ont pour objectif de figer les dispositions qui doivent être comprises dans les CPER. La commission émet donc un avis défavorable.

et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie. Le Gouvernement s'engage ainsi à privilégier, en zone dense, les investissements permettant la réduction de l'usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion et accompagnera les collectivités dans leurs projets.

pertinents. En matière de moyens, l'État prévoit 1,1 milliard d'euros d'ici à 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien.

Le présent amendement tend donc à fixer à 200 millions d'euros par an le montant des appels à projets. Cet investissement est indispensable pour augmenter les retombées économiques directes du vélo, qui représentent déjà 4,5 milliards d'euros en France et qui pourraient aisément être décuplées si un investissement suffisant permettait de faire croître l'usage de ce mode de transport. On estime à 5,6 milliards d'euros par an le bénéfice en matière de santé des 4,6 milliards de kilomètres parcourus annuellement à vélo.

Madame la ministre,

De plus, le train est plus que jamais un moyen de locomotion d'avenir : comme les milieux urbains, les territoires ruraux aspirent à développer les transports collectifs pour limiter l'utilisation des voitures, afin de préserver l'environnement. Qu'elles soient utilisées ou pas, les lignes de chemin de fer en zone rurale doivent être préservées, car de nouvelles technologies et techniques de transport sur voies ferrées, moins polluantes- leur bilan carbone est neutre -, moins lourdes pour la structure de voie, plus souples dans le cadencement et la gestion des passagers et plus économiques sont en passe de voir le jour.

pourrait voir le jour industriellement d'ici à 2023. En conséquence de ces développements prochains, et compte tenu de la volonté des collectivités locales concernées, les lignes aujourd'hui désaffectées et leurs emprises doivent être préservées

Je vous rappelle que le Gouvernement a assigné à la France l'objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour cela, il est nécessaire que le système énergétique évolue afin que les énergies consommées sur le territoire français n'émettent plus de gaz à effet de serre. Stocker l'hydrogène permettrait de stocker des énergies renouvelables, ce qui constituerait une avancée majeure dans la transition écologique et solidaire annoncée et largement attendue. Outre la transition écologique, promouvoir la filière hydrogène offrirait une possibilité de reconversion importante et crédible à notre économie et à nos usines. Promouvoir l'hydrogène permettrait à notre pays de rattraper son retard en la matière. Dans un rapport publié l'année dernière, le cabinet McKinsey soulignait que la filière de l'hydrogène pourrait atteindre 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représenter plus de 150 000 emplois.

n'est pas financé par l'Afitf. Sous cette réserve, et dès lors qu'il est bien compris par tout le monde que nous ne mettons pas à la charge de l'Afitf des investissements qui sont, à l'heure actuelle, soutenus par d'autres dispositifs, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée.

rappelle que la France et l'Allemagne sont actuellement leaders dans ce secteur en matière de recherche et développement. Si nous n'y consacrons pas les moyens appropriés, nous serons très vite dépassés, en particulier par la Chine. Il serait regrettable que nos savoir-faire ne nous permettent pas

C'est une manière de s'assurer que les projets de mobilité tiennent compte du végétal et que les infrastructures vertes soient envisagées comme des réponses essentielles pour relever les défis environnementaux et urbains actuels.

? Je soutiens naturellement la biodiversité en général et la végétalisation des infrastructures en particulier, mais il me semble que, s'il s'agit d'une ambition louable, l'introduction d'une obligation généralisée de végétalisation des infrastructures de mobilité

le réseau d'infrastructures existant et notamment la complémentarité offerte par le transport fluvial et le transport maritime. Il vise également à faire entrer les marchandises en zone urbaine, à permettre la mise en oeuvre de logistiques massifiées au coeur des agglomérations